La séance est ouverte.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. La parole est à Mme Valérie Létard, pour un rappel au règlement. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 42 de notre règlement. Elle concerne l'organisation de nos débats et la considération que le Gouvernement porte à nos travaux. Texte après texte, projet de loi après projet de loi, nous ne pouvons que constater l'absence d'intérêt manifesté par le Gouvernement pour les propositions et les apports du Sénat, que ce soit en commission ou en séance publique. Le groupe Union Centriste s'indigne de cette situation et souhaite que le Gouvernement revienne à la raison. En matière de logement, le Sénat, grâce à son président, Gérard Larcher, a organisé la conférence de consensus dès la fin de l'année dernière. Après les annonces brutales du Gouvernement sur le financement du logement social, nous avons tous décidé d'aborder le texte portant évolution du logement, de l'aménagement pas été perçu puisque le Gouvernement a choisi de saisir, comme à chaque fois, l'Assemblée nationale en première lecture, mais désormais le traitement dont fait l'objet le Sénat n'est pas amélioré. Chaque groupe politique a travaillé. La commission des affaires économiques et sa rapporteur ont établi il y a deux semaines un texte de loi dont nous examinons le contenu dès aujourd'hui. Cette nuit, le Gouvernement a déposé de nouveaux amendements, venant s'ajouter à de nombreux autres et visant notamment à revenir à la rédaction initiale de son texte et à balayer le travail du Sénat, avant même d'en avoir débattu.

Quel sera le sort de nos avancées ? Comment travailler sérieusement et utilement si le Gouvernement ne respecte ni nos calendriers ni nos propositions ? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire dans quelle direction nous devons aller avec vous ? Car c'est bien ce que nous voulons : aller avec vous, mais en direction de l'intérêt de nos concitoyens, et d'une politique territoriale équilibrée et juste.

les méthodes employées par le Gouvernement sont indignes de la démocratie. Nous vivons une session dite « extraordinaire », qui se transforme finalement en un déferlement soudain de textes législatifs tous plus importants les uns que les autres, qui visent à transformer en profondeur la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens et l'organisation même de nos territoires. Monsieur le ministre, répondez-nous

au cours de ma vie parlementaire, et même avant, j'ai toujours eu une considération particulière pour la représentation nationale et pour le bicamérisme.

tant d'estime. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

n'est pas une vanité stylistique qui viendrait, à un moment, esthétiser un acte de construire, même si cette fonction esthétique, on le sait, est l'une de ses facettes évidentes. Loin d'être superflue, elle est tout simplement essentielle à la collectivité, au mieux vivre ensemble, et donc à nos concitoyens.

l'architecture n'est plus un enjeu purement technique laissé aux spécialistes et aux artistes du bien construire. Elle est devenue un enjeu collectif, un enjeu civique, que chacun peut s'approprier en tant que citoyen.

car elle est à la confluence de nombreux défis : l'aménagement du territoire, la qualité de la construction, la question écologique, la réduction de la dépense énergétique, mais aussi la question civique de la mixité sociale et celle du bien être ensemble. En d'autres termes, et nous le savons, mes chers collègues, l'architecture est porteuse de représentations, tout comme le sera le patrimoine. Elle conditionne ce que nous pouvons faire, elle impacte notre manière de vivre, mais atteint aussi ce que nous sommes. Alors oui, par-delà la conception esthétique, elle est vraiment l'expression d'une vision de la cité dans un espace donné. La transformation que connaissent nos villes, nos territoires, particulièrement sous l'influence du numérique, rend encore plus impérieux le travail effectué par ces penseurs d'espace, par ces modélisateurs du monde. Quels bâtiments voulons-nous demain ? Comment construire ? Comment développer une ville et un territoire intelligents ? Comment améliorer le cadre de vie quotidien de nos concitoyens ? Telles sont les problématiques qui fondent toute réflexion sur l'architecture. En tant que représentants des collectivités territoriales, nous ne pouvons y être que sensibles.

En effet, par la création de ces nouveaux outils que sont les projets partenariaux d'aménagement, les PPA, et la grande opération d'urbanisme, la GOU, il s'agissait- rien de moins ! -que de retirer aux communes la maîtrise de leur aménagement, puisque de telles opérations auraient pu voir le jour en dépit de la volonté des communes. ces mêmes communes n'auraient plus disposé de compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, du fait d'un mécanisme de transfert automatique. Cet article, sous couvert de partenariat collectivité-État, renforçait ainsi dangereusement le processus de transfert des compétences des communes vers les intercommunalités, notamment en matière d'urbanisme, et confirmait ainsi la volonté de faire des communes des coquilles vides. Que l'État dispose de prérogatives particulières dans le cadre des opérations d'intérêt national, cela relève de la légitimité de la puissance publique ; mais que les intercommunalités puissent imposer des projets aux communes, nous ne le souhaitons pas. La commission des affaires économiques, sous l'impulsion de Mme la rapporteur, et à la suite des amendements que nous avons déposés, a significativement modifié cet article en renforçant la place des communes. Ainsi, la commune est dorénavant signataire de droit d'un PPA et elle pourra s'opposer au transfert de compétence concernant les autorisations d'urbanisme. C'est une bonne chose, même si nous proposons d'aller encore plus loin, notamment en rendant non seulement de droit mais également incontournable la signature de la commune, en tant que signe de son accord avec ce projet. Nous estimons, en effet, que rien ne doit pouvoir se faire sans l'accord de la collectivité de base, cet échelon démocratique qu'est la commune. Il n'en reste pas moins qu'à nos yeux ce processus partenarial s'insère dans une vision très centralisatrice de l'aménagement, une vision qui ne fait pas confiance aux territoires et aux élus pour mener les politiques utiles aux habitants et répondant aux enjeux de transports, de logement, de développement économique. Que l'État soutienne les collectivités territoriales, c'est une chose, mais qu'il impose sa vision de l'aménagement, c'en est une autre,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi, en préambule, de livrer quelques données chiffrées et informations concernant l'habitat en Martinique. Notre île se caractérise par une faible mobilité résidentielle : les deux tiers des ménages habitent dans le même logement depuis plus de huit ans, contre 62 % en Guadeloupe et 57 % en France hexagonale. Les prix élevés de l'immobilier limitent l'accession à la propriété, malgré le fort désir de devenir propriétaire chez les ménages martiniquais. Les ménages les plus jeunes et les plus modestes sont toujours en situation de surpeuplement. Le loyer moyen au mètre carré dans le parc privé est plus onéreux en Martinique qu'en Guadeloupe et dans l'Hexagone. Enfin, la croissance du parc de logements martiniquais est réelle, mais insuffisante. C'est pourquoi ce projet de loi aurait pu présenter un intérêt certain pour nos territoires. Or nous ne sommes que peu concernés, en l'état actuel des choses, par ce texte. En effet, comment un texte prétendant vouloir « construire plus, mieux et moins cher » peut-il ne contenir aucune disposition relative au concept de résilience quant aux politiques publiques de l'habitat ? De la même manière, je suis de ceux qui promeuvent une approche plus territorialisée des politiques du logement, qui tendrait vers « une nouvelle gouvernance publique et une meilleure adéquation avec les réalités locales », dans la mesure où il existe une forte différenciation entre ces dernières. Les approches horizontales favorisant les coopérations et les mutualisations locales ont autant de pertinence que les approches verticales et budgétaires. Ainsi, l'évolution des organismes de logement social doit leur permettre, à terme, de conduire leurs actions en cohérence avec les politiques menées par les collectivités locales, les métropoles ou les départements de leurs lieux d'intervention. Tout cela me conduit à dire que ce texte est loin d'être parfait. C'est pourquoi j'ai proposé un certain nombre d'amendements allant dans le sens de l'intérêt de nos territoires. La parole est à Mme Michelle Gréaume, Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières années, nous avons constaté une volonté centralisatrice dans les politiques d'aménagement, volonté qui rompt avec l'esprit des lois de décentralisation de 1983. En effet, depuis cette date, les communes disposent de la compétence de principe en matière d'aménagement, et du pouvoir d'autorisation en matière de droit des sols. C'est une bonne chose et ce principe ne doit pas être remis en question. L'État dispose déjà du droit, s'il existe des projets spécifiques répondant à des enjeux particuliers d'intérêt général, d'arrêter une opération d'intérêt national, une OIN. Nous considérons que cette faculté doit être utilisée sans avoir recours à d'autres procédés. Car au fond, avec cet article, derrière l'affichage de partenariat, c'est bien cette volonté centralisatrice qui s'exprime, tout comme celle visant à faire de l'intercommunalité l'interlocuteur unique sur un territoire. Nous sommes donc particulièrement satisfaits d'avoir été entendus en commission sur le rôle central du maire et de la commune comme cellule de base de la démocratie. Mme la rapporteur a porté avec nous des amendements en ce sens, et nous estimons que l'évolution de ce texte est largement favorable. Nous considérons en effet que les élus locaux, je dirai même communaux, ne peuvent être sortis de la boucle des projets d'aménagement, qui ne peuvent se concevoir sans l'accord des territoires concernés au plus près des réalités de terrain. Un bon projet, c'est un projet accepté, dialogué, travaillé en intelligence entre tous les échelons, avec tous les partenaires, de l'État à la commune, sans oublier la population. C'est cette conception de la démocratie locale que nous portons et que nous avons voulu traduire au travers de nos amendements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Avec cet amendement, nous souhaitons aller dans le sens des travaux menés en commission, lesquels ont rendu obligatoire l'accord de la commune pour les grandes opérations d'urbanisme. Nous voulons

indispensable et incontournable pour permettre l'existence même du projet partenarial, support des grandes opérations d'aménagement. Nous demandons donc, comme une formalisation de l'accord de la commune, que sa signature soit obligatoire et non de droit. C'est une

NOTRe ... Le maire doit pouvoir justifier auprès de ses concitoyens des projets d'aménagement sur son territoire. Il est donc normal qu'il soit signataire de tout contrat ou projet dont l'assise est le territoire communal. C'est la base même de notre démocratie. Quel est l'avis de la commission

Il permet simplement aux parties de s'accorder sur les grandes lignes de l'aménagement. Je vous rappelle également que les communes qui le désirent sont signataires de droit d'un PPA, en vertu du texte qui a été adopté par la commission.

dispose seule de la légitimité démocratique pour l'aménagement d'un territoire. Que des personnes privées soient intéressées, par exemple, par de grandes opérations d'urbanisme, c'est une chose ; c'en est une autre de leur permettre d'être signataires de ce contrat. Nous estimons donc qu'il convient de recentrer la signature de ce projet sur les personnes publiques, qui représentent l'intérêt général. Quel est l'avis de la commission

rapporteur de la commission des affaires économiques est parfaitement claire et elle a le mérite de la lisibilité, mais l'amendement de la commission des lois tend à replacer les communes au centre du dispositif tout en se prémunissant contre d'éventuels risques de blocage. Pour avoir quelque expérience en la matière, je crains que, si

qui, de la commune ou de l'EPCI, se prononcera sur le permis de construire ou sur le permis d'aménager. Par ailleurs, tout transfert de compétence vers l'échelon intercommunal

que tout transfert de compétence à l'EPCI devra impérativement recueillir l'avis conforme des maires. Lorsqu'un maire sera consulté sur la création d'une GOU, il devra préciser

Ce n'est pas moi qui ai voté la fusion obligatoire des régions. Moi non plus ! Ce n'est pas moi qui ai voté la loi NOTRe

et en aura précisé le périmètre et les caractéristiques. Dès lors, pourquoi le projet de loi prévoirait-il que l'État donne son accord préalablement au lancement de la GOU ?

Au regard de ce constat, la création, ces dernières années, des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPENAF, a permis la mise en place de projets urbains plus économes en espaces agricoles et naturels, un dialogue renforcé entre les différents acteurs de l'aménagement. où il est vital de rendre nos territoires résilients, l'application, en amont des projets, d'une logique d'aménagement fondée sur le principe d'évitement et de réduction est seule garante de la pérennisation du capital représenté par les espaces agricoles et naturels.

ni d'une autorisation d'urbanisme. Dans ce cadre, je ne vois pas pourquoi la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers disposerait d'éléments plus précis pour se prononcer. Il ne paraît pas justifié de requérir son avis au moment de la délimitation du périmètre de la GOU. Par conséquent, la

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la possibilité, pour le préfet, de passer outre l'avis défavorable d'une commune, afin de permettre à la collectivité territoriale

Cet amendement vise à rétablir l'obligation de faire figurer le montant de la participation due au titre des équipements propres dans l'autorisation ou la déclaration d'urbanisme. Il procède du même esprit que la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural

: La parole est à M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à reconnaître la pluridisciplinarité réelle des intervenants dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement, au bénéfice des maîtres d'ouvrage. Chacun le sait, les opérations d'aménagement et de lotissement nécessitent de recourir à des compétences pluridisciplinaires. Selon les sites et la nature des projets, certaines compétences peuvent être prépondérantes, telles que la capacité à assumer la composition et l'ordonnancement général de l'opération ou à prendre en compte la biodiversité, l'aspect environnemental,

disposent tous, sur le plan de la maîtrise d'oeuvre, des assurances nécessaires en cas de faute avérée. Il n'y a donc ni problème de compétence ni difficulté administrative particulière pour qu'ils puissent intervenir en toute sécurité pour un ordonnateur public ou privé. Le maître d'ouvrage

de définir une démarche cohérente et son contenu, il ne lui revient pas de fixer un cadre si étroit de réalisation ni surtout de réserver des opérations à certains corps de métier en en excluant d'autres, dès lors que tous disposent des compétences et des capacités administratives suffisantes.

L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme précise que la demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage. C'est pourquoi tous les professionnels compétents pour établir un PAPE,tels que les architectes, au sens de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les paysagistes concepteurs, au sens de l'article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les géomètres-experts, au sens de l'article 1de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, doivent pouvoir accompagner le porteur d'une demande de permis d'aménager pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret.

une meilleure qualité des cadres de vie. Cet amendement a pour objet de réintroduire en le complétant l'article 1, afin de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l'exigence de pluridisciplinarité dans l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental

L'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental nécessaire à l'obtention d'un permis d'aménager préalable aux projets de lotissement exige un travail d'équipe pluridisciplinaire, mettant en oeuvre des compétences complémentaires.

1dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, afin de permettre aux paysagistes concepteurs d'être mandatés au même titre que les architectes en vue de l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental accompagnant la demande de permis d'aménager.

libre choix de l'aménageur. Seul le recours à l'architecte est obligatoire. Il permet en effet de garantir la bonne intégration paysagère des grands projets de lotissement, qui peuvent, de fait, avoir un fort impact environnemental et paysager. Il me semble que

à un architecte ou à un paysagiste concepteur. La commission de la culture a débattu du sujet et a estimé qu'il fallait laisser l'architecte au coeur du projet d'aménagement.

établissant la division foncière. Il identifie en particulier les espaces collectifs et les voiries, à l'aide de plans de masse, de photographies, d'éléments de topographie. En tant que professionnels concourant à l'aménagement du cadre de vie, tant les architectes que les paysagistes concepteurs les compétences requises pour élaborer un PAPE. Il est dès lors souhaitable, afin de promouvoir la qualité urbaine des lotissements, de permettre aux porteurs de projet de recourir, au choix,

évoqué des équipes pluridisciplinaires : il est en effet important de conjuguer les avis pour faire en sorte que le monde soit beau. Maires ou anciens maires, nous avons besoin de donner de la couleur à la vie, à nos paysages.

et les régions, en matière de gestion des espaces naturels sensibles, de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, de politiques de solidarité, pour les premiers, de programmation, de planification et d'encadrement de l'action des collectivités, de définition des orientations en matière de développement

L'équivalent d'un département disparaît tous les sept ans du fait de l'urbanisation. Une telle situation ne peut perdurer. Il convient de créer les garde-fous nécessaires pour s'assurer que cette urbanisation répond bien à un motif d'intérêt général et vérifier que des alternatives moins consommatrices de terres agricoles ne sont pas envisageables. Au regard de ce constat, nous estimons pertinent de soumettre à un avis conforme, et non à un avis simple, de la commission départementale de préservation des espaces naturels,

a pour mission de gérer le patrimoine foncier agricole en lui redonnant sa valeur d'outil de travail, de permettre le développement et les mutations de l'agriculture, ainsi que l'installation de nouveaux agriculteurs, d'éviter le mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers, de préserver les paysages et la biodiversité, de lutter contre l'érosion des sols et de protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques. Ces missions sont fondamentales pour la préservation des richesses naturelles des territoires d'outre-mer. Aussi, pour les grands projets d'envergure, il est plus prudent de renforcer, dans les régions d'outre-mer, le caractère obligatoire de l'accord de la CDPENAF,

fortement le paysage urbain de certains territoires. Elles doivent donc être exemplaires de tout point de vue, qu'il s'agisse du respect des procédures de participation du public, des procédures d'urbanisme ou des règles d'attribution des marchés publics, afin d'en garantir la qualité architecturale, urbaine et environnementale. La réalisation de tout type d'équipement public, bâtiment ou infrastructure dans leur périmètre doit donc relever des principes imposés par la loi MOP de 1985, qui fixe le cadre relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et de ses rapports avec la maîtrise Cette loi permet principalement la reconnaissance du principe de séparation juridique et fonctionnelle entre le maître d'ouvrage public, qui définit et commande, le maître d'oeuvre, qui conçoit et dirige, et l'entreprise qui exécute. Ces règles ont permis de maintenir la qualité architecturale du bâti, sa durabilité et son caractère innovant. Elles ont également servi à éviter de nombreuses malfaçons liées à la volonté du moindre coût de réalisation et, par conséquent, des surcoûts supplémentaires. Cet équilibre doit être respecté au sein des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme, sauf à vouloir des équipements publics de faible qualité, non durables et qui représenteront à terme un coût plus important pour la collectivité. Nous proposons donc de supprimer la dérogation prévue dans cet article à la loi MOP, qui va dans le sens d'une technocratisation à outrance de l'aménagement et de la construction. La parole

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures de dérogation à la loi MOP, qui aboutissent progressivement à la vider de son contenu. Ce n'est pas la bonne méthode ! La loi MOP pose les principes généraux de la maîtrise d'ouvrage publique et de ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre. La qualité et la maîtrise financière d'une opération tiennent pour une part importante à la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.

ouvrages d'infrastructures situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ou d'une grande opération d'urbanisme- autant dire que l'on ne parle pas de petites infrastructures ! Il semble

de préservation de l'environnement et du cadre de vie et de qualité architecturale et urbaine dans le cadre contractuel du projet partenarial d'aménagement et, le cas échéant, des traités de concession d'aménagement conclus avec les aménageurs. Le Gouvernement

le type de normes qui seront concernées, dans le cadre du décret à venir, par la mesure que nous allons voter.

identifie précisément les règles auxquelles il est dérogé. Le projet de loi prévoit que ces dérogations font l'objet d'une étude de faisabilité et de résultats validée par l'établissement public d'aménagement ou par le préfet. La loi et l'autorité administrative encadrent déjà fortement ce dispositif, tout en permettant aux maîtres d'ouvrage de proposer et de justifier eux-mêmes les dérogations demandées. Il n'est pas judicieux de les encadrer davantage par décret. La commission émet

Nous sommes donc hostiles à ce que s'applique aux opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté une procédure de participation du public dérogatoire au droit commun, qui fasse l'impasse sur une enquête publique en bonne et due forme. Nous sommes également opposés à ce que l'ouverture et l'organisation de la participation du public par voie de participation électronique fassent partie des compétences que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. Cela n'a l'air de rien, mais, de loi en loi, on rabote la participation du public au nom de l'efficacité et de la rapidité. Nous considérons, bien au contraire, qu'il s'agit d'un temps utile et nécessaire, celui de la démocratie, pour améliorer les projets et construire

sont très présents dans l'action que je mène. Étant issu d'un territoire où la desserte internet est particulièrement difficile, je suis préoccupé par ces problèmes,

obligatoire. Selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, ces procédures ne relèvent pas du dispositif de concertation préalable du code de l'urbanisme, reposant notamment sur l'exercice du droit d'initiative. les procédures de mise en compatibilité du SCOT et du PLU, ainsi que l'élaboration et la révision des cartes communales entrent bien dans le champ de la concertation préalable du code de l'environnement, dès lors qu'elles sont soumises à une évaluation environnementale. Ce double régime est source de complexité et d'insécurité juridique pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à soumettre ces deux dernières procédures à la concertation obligatoire prévue par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. Ses auteurs visent ainsi un double objectif : la simplification du régime de participation du public applicable aux documents d'urbanisme et

et révisions des SCOT et PLU, alors que les autres procédures d'évolution des SCOT et des PLU relèvent de la concertation du code de l'environnement. Certains jugent peut-être que cette distinction est

Gontard, sur l'article. Le présent article ambitionne de simplifier un certain nombre de dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté et aux concessions d'aménagement. Si certaines de ces mesures ne présentent pas de difficulté particulière, ce premier coup de canif porté à la loi MOP nous inquiète grandement. Ainsi, c'est un autre outil à la disposition des communes, à savoir les concessions d'aménagement, qui pourrait ne plus relever demain du code des marchés publics et du champ d'application de la maîtrise d'ouvrage publique. Les exceptions à la loi MOP sont très rares et doivent le rester. Si elle mérite sans doute quelques aménagements, notamment pour une meilleure prise en compte de la performance énergétique des bâtiments, cette loi satisfait l'ensemble des acteurs du secteur et doit demeurer la colonne vertébrale de la commande publique et de la construction dans notre pays.

Elle permet à tous nos artisans locaux- peintres, électriciens, plombiers, maçons ... -, de bénéficier de la commande publique et de pouvoir compter sur une activité pérenne. Chaque fois que l'on contourne la loi MOP par des dispositifs de type conception-réalisation, l'on privilégie les grands groupes au détriment des TPE de nos territoires.

très précis et permet de clarifier les missions des intervenants. La construction et la commande publiques ont évolué ces dernières décennies, sous l'influence de la législation européenne. Certes, cette loi aurait sans doute nécessité d'être actualisée pour fluidifier les liens entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, simplifier des procédures ou s'adapter aux enjeux modernes que constituent la protection de l'environnement et la maîtrise énergétique. Ce que nous trouvons dommage, c'est que le Gouvernement ait préféré suivre une autre voie

objectifs à valeur constitutionnelle, et elle ne va pas dans le sens d'une plus grande sécurité juridique, finalité partagée par les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage, eu égard aux lourdes problématiques que soulèvent les contentieux. La preuve que la loi MOP constitue un frein au bien construire n'a, me semble-t-il, pas été pleinement apportée.

Or les projets réalisés dans le cadre d'une ZAC sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement. Pour autant, d'après le droit en vigueur, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement

Afin de conforter la notion de projet d'ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, le présent amendement vise à prévoir les projets composant d'une ZAC en amont, en rassemblant les concertations préalables de ces projets composantes sous le « chapeau » de la participation du public prévue pour le projet d'ensemble mené sous forme de ZAC. Cependant, il convient de préciser que les projets composant la ZAC, non intégrés lors de la concertation de la ZAC, demeurent soumis à la concertation prévue à l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement. Quel est l'avis de la commission

donc un avis favorable sur cet excellent amendement, présenté par votre excellent collègue

Quelle est la situation actuelle ? La procédure de création d'une ZAC dans le cadre d'un projet d'aménagement est soumise à une concertation préalable obligatoire au titre du code de l'urbanisme. Elle est exemptée de concertation préalable au titre du code de l'environnement.

permet qu'un projet d'ensemble soit soumis à une seule concertation préalable obligatoire en amont au moment de la concertation sur création de la ZAC. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir deux concertations

Ce sont des opérations d'envergure, dont les enjeux sont importants. Les bâtiments publics à réaliser doivent relever des principes de la loi MOP, qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d'ouvrage publics qu'aux prestataires privés. La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d'une opération d'aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP. Cela évite tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l'argent public.

aux grosses sociétés, qui ne sont pas dans l'écoute et qui sont, souvent, à l'origine de contentieux. La majorité gouvernementale souhaite supprimer l'intervention des architectes dans les opérations des projets d'envergure. Nos grands architectes iront embellir d'autres pays que la France ! Sans architecte, nous n'aurions eu ni Beaubourg, ni la Grande-Motte, ni la pyramide du Louvre ! On aurait pu s'en passer ... Sans nouveaux rêves, la France sera le pays d'un patrimoine sans avenir

qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d'ouvrage publics qu'aux prestataires privés, les objectifs étant l'intérêt général et la protection des usagers finaux. Les alinéas 23 et 24 de l'article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi la voie d'une concession d'aménagement de réaliser des bâtiments publics avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP. loi MOP. Avec ces nouvelles dispositions, les bâtiments publics situés dans le périmètre d'une opération d'aménagement ne seront plus tenus de respecter les règles de passation des marchés publics. La qualité architecturale des constructions sera laissée au bon vouloir de l'aménageur, ce dernier n'étant tenu qu'à une obligation de surface de construction à produire. La contrainte administrative liée à l'organisation des procédures MOP pourrait être bientôt jugée insurmontable par les communes moyennes, au regard de la simplicité d'une convention d'aménagement. Pourtant, la qualité de nos villes, leur lisibilité, le sentiment de bien-être qui y règne sont conditionnés par la différentiation des fonctions et la variété des espaces. La construction pertinente de la ville ne peut pas se limiter à la réalisation des voiries et des réseaux. la qualité des constructions publiques est le premier vecteur de réussite d'un nouveau quartier ou d'une rénovation urbaine. La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d'une opération d'aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l'argent public.

supprimer les dispositions du projet de loi rendant plus opérationnelle la convention de participation des constructeurs au financement des équipements publics en ZAC. Les deux amendements ne se réfèrent

très clairement au Sénat qu'il ne s'agit aucunement de supprimer le recours aux architectes. Dans ma vie précédente, j'ai pu constater que les avocats étaient beaucoup moins forts pour se défendre que les architectes

crée un nouveau cas de dérogation à la loi MOP, permettant à l'aménageur qui passe par la voie d'une concession d'aménagement de réaliser des bâtiments publics avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.

relever de la loi MOP. L'argent public est denrée suffisamment rare aujourd'hui. Il faut l'utiliser avec précaution et à bon escient ; on ne cesse de nous le répéter ... Le respect de la loi MOP impose une démarche de qualité tant aux maîtres d'ouvrage publics qu'aux prestataires privés, l'objectif étant bien l'intérêt général. Dédouaner les collectivités du respect de cette loi MOP ouvre la voie à un changement drastique des règles de construction, de l'exigence de qualité du bâti, de la durabilité

supprimer la disposition du projet de loi qui exclut du champ de la loi MOP tous les ouvrages ou bâtiments réalisés par des aménageurs intervenant dans le cadre d'une concession d'aménagement.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, un maître d'ouvrage public peut procéder soit en régie directe pour faire son opération d'aménagement, soit par mandat, soit par concession. Mais il est prévu que le concessionnaire puisse être privé puisse être privé ou public. Cette disposition s'applique à tous les concessionnaires, qu'ils soient publics ou privés. Rien ne justifie qu'un aménageur public logiquement soumis aux dispositions de la loi en tant que maître d'ouvrage public n'y soit plus soumis. soumis. Les aménageurs privés ne sont déjà pas soumis aux dispositions de la loi MOP lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une concession d'aménagement ; le recours à ce type de contrat se traduit par un transfert de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale vers l'aménageur.

s'applique sur l'ensemble du territoire en l'absence de circonstances ou de zones déterminées à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiments réalisés dans le cadre d'un contrat de concession

elle détermine le rôle et les missions du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre par rapport à la construction envisagée. D'autre part, elle permet aux entreprises de disposer de plans, de quantitatifs et d'études d'exécution pour réaliser leur offre technique et de prix. loi rationalise également les documents préparés en amont de la consultation, en vue d'une réponse précise des entreprises. L'étude fine des besoins et de qualité en amont contribue à bien prévoir les travaux nécessaires et à limiter les avenants en cours d'exécution des travaux. Toutes les entreprises répondent alors selon les pièces précitées. Cela permet au maître d'ouvrage de comparer plus facilement les offres des entreprises. Cela évite à chaque entreprise de consulter un bureau d'études en amont, donc d'engager des frais sans avoir la certitude à ce stade de remporter le marché. C'est un réel levier pour l'accès direct des TPE aux marchés publics. Cela permet à la concurrence de s'exercer dans des conditions saines et aux entreprises de disposer en amont de plans estimatifs, quantitatifs et études d'exécution. Les entreprises pourraient ainsi remettre leur offre technique de qualité à des prix maîtrisés, de nature à respecter les cadrages budgétaires. La dérogation envisagée dans le présent article semble disproportionnée. Elle s'appliquerait à l'ensemble des concessionnaires d'une opération d'aménagement, quelle que soit leur nature, privée ou publique.

et du mandat. Il semble toutefois que cette disposition crée une très large dérogation à la loi MOP, dans les cas où le concessionnaire est, lui aussi, maître d'ouvrage

un problème et s'interroge sur le régime juridique dans lequel elle doit se placer pour les bâtiments qu'elle veut faire réaliser : soit c'est celui de la concession, au même titre que les autres travaux et équipements concourants à l'opération, soit c'est celui de la loi MOP. La disposition introduite La disposition introduite dans le projet de loi, au contraire, vise à sécuriser l'action de la collectivité en soumettant clairement tous les éléments de l'opération d'aménagement- travaux, équipements, bâtiments -au seul cadre juridique de la concession d'aménagement lorsque

aux maîtres d'ouvrage de faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre, architectes et bureaux d'études, en un seul bloc, alors qu'il est effectivement possible de réaliser un certain nombre d'économies. C'est ce que nous disent, sur le terrain, non seulement

: je le répète, cet équilibre qui avait été trouvé dans les textes s'est transformé sur le terrain. Il ne me semble pas souhaitable que, une fois de plus,

demande expresse de l'Union européenne -à retrouver la règle de l'allotissement dans des conditions optimales. Cet équilibre ayant été atteint, il ne faut pas le démolir. La parole est

l'idée de la suppression des alinéas 29 et 30 portée par un certain nombre de collègues, dont le rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. L'ensemble

un projet, plan ou programme à évaluation environnementale, dans le cadre de l'examen au cas par cas, précise les objectifs spécifiques de cette dernière. Il ne nous semble ni réaliste ni efficace de systématiser à ce stade de la décision une telle évaluation. Cela pourrait être source de complexité et alourdir la décision d'examen au cas par cas, les délais de l'ensemble des dossiers risquant d'être affectés et les cadrages insuffisamment contextualisés, donc peu pertinents. Il convient, à notre sens, de valoriser le dialogue, sur l'initiative du porteur de projet, plan ou programme. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à supprimer les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale.

est à M. le ministre. Par cet amendement, nous voulons ouvrir la possibilité de recourir à la procédure de réquisition temporaire pour l'organisation et le déroulement des jeux de Paris de 2024.

Jeux de 2024. La loi autorise déjà le recours à la procédure d'expropriation en extrême urgence pour cause d'utilité publique prévue par le code de l'expropriation. Quand il s'agit des jeux Olympiques, les dérogations sont beaucoup plus faciles. Le présent amendement vise à reprendre les préconisations du rapport de l'Inspection générale des finances du 30 mars dernier, qui recommandait la mise en place de ce dispositif pour pallier, le cas échéant, les difficultés éventuelles, en permettant une action plus proportionnée aux nécessités des jeux Olympiques et plus respectueuse des droits des citoyens. Une disposition similaire de réquisition temporaire avait été prévue à l'occasion des jeux Olympiques d'Albertville et de Savoie par la loi du 31 décembre 1987. Notre amendement vise à la reprendre et à l'élargir, compte tenu de la topologie des lieux concernés. Il a également pour objet de reprendre les dispositions protectrices essentielles, à savoir l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation et la remise en état avant restitution aux bénéficiaires de la réquisition.

de l'expertiser. Sur le principe, il semble préférable, quand cela est possible, de privilégier la réquisition temporaire à l'expropriation.

d'expropriation, qui serait moins attentatoire au droit de propriété. Nous pensons, à l'opposé, que la réquisition temporaire est plus attentatoire au droit de propriété.

Une personne ou une entreprise est expropriée. Elle recevra une juste et préalable indemnité correspondant à la valeur vénale de son bien et elle pourra se réinstaller ailleurs. Une personne est réquisitionnée temporairement. Elle recevra une indemnité qui couvrira seulement sa privation de jouissance.

En début de séance, deux sénatrices ont à juste titre effectué un rappel au règlement pour dénoncer des méthodes légistiques qui n'en sont pas. Pourtant, lors de la révision constitutionnelle, on ne manquera sans doute pas de nous faire la leçon sur la meilleure façon de fabriquer la loi

mais je pense que le Parlement, dans son ensemble, a atteint la limite de l'exercice. Une conférence des présidents se tiendra

doit mentionner son bénéficiaire, préciser l'usage pour lequel celle-ci est ordonnée, opérer le transfert du droit d'usage et autoriser le bénéficiaire à prendre possession.

quant à la réalisation des équipements dans les enveloppes et les délais impartis. Il se trouve qu'une mission conjointe de l'Inspection générale des finances, de la jeunesse et des sports et du développement durable

adopté une vision plutôt positive de ce projet de loi, pour faire en sorte que les jeux Olympiques se passent le mieux possible, et nous avions donné au Gouvernement les moyens juridiques d'organiser les jeux Olympiques dans les meilleures conditions. Il me semble que c'est encore ce que nous demande le Gouvernement aujourd'hui,

concerne les nominations au comité consultatif de l'établissement Paris-Saclay. Comme vous le savez, mes chers collègues, entre la brutale interruption de l'exposition universelle

a prévu la mise en compatibilité accélérée et simplifiée des documents d'urbanisme, pour permettre la réalisation dans les temps des constructions et opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques. Cet article est également applicable aux constructions et opérations qui ne contiennent que que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique. Or certaines constructions ou opérations contigües à des sites nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux, déjà engagées programmées à ce jour, pourraient affecter les conditions de desserte, d'accès, de sécurité ou d'exploitation de ces sites si elles ne sont pas achevées d'ici à 2024. Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice des dispositions de l'article 12 à ces constructions et opérations d'aménagement contigües, dont il est précisé que la liste sera fixée par décret. Au vu des circonstances exceptionnelles que constitue l'organisation des jeux Olympiques en 2024, il est judicieux de faire bénéficier ces opérations périphériques de procédures simplifiées, en adaptant les procédures d'urbanisme et en recueillant les participations du public.

Or, dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d'inscrire l'investissement dans son budget. L'inscription dans le programme des équipements publics permet d'assurer la réalisation et le financement d'un équipement public dans le cadre d'une opération d'ensemble. De plus, en retour, l'équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession. L'accès des projets réalisés dans le cadre d'opérations d'aménagement aux subventions de la DETR permettra d'en accélérer la réalisation sur l'ensemble des territoires ruraux. Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l'article L. 2334-33 du CGCT pour permettre le financement d'équipements publics d'intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d'une concession d'aménagement confiée à une société publique locale, une société d'économie mixte locale ou une société d'économie mixte à opération unique.

Gouvernement ? Aujourd'hui, en l'état du droit, les concessionnaires d'aménagements ne figurent pas dans la liste limitative des bénéficiaires de la DETR, c'est exact.

aux dotations budgétaires qui sont réservées aux collectivités locales et aux EPCI. L'attribution directe d'une part de DETR à une entreprise être qualifiée d'aide d'État au sens du droit européen, ce qui supposerait une analyse spécifique, tout nouveau régime d'aide devant être notifié à la Commission européenne.

Il s'agit d'un amendement de coordination. La rédaction du second alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d'aménagement. D'une part, l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme définit tant la notion d'aménagement que celle d'opération d'aménagement. Or ces définitions dépassent par leurs implications et leurs applications le seul livre III du code de l'urbanisme dédié à l'aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l'aménagement. D'autre part, la référence à ce seul livre à l'article L. 300-1 n'apparaît pas totalement compatible avec le premier alinéa de l'article L. 300-4 du même code, qui fait clairement référence aux « opérations d'aménagement prévues par le présent code ». La notion d'aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC. Cette référence n'est pas sans impact sur le champ d'activité des sociétés publiques locales, outil de coopération publique-privée né d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale adoptée à l'unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010. Cette rédaction est plus limitative que celle qui pour les sociétés publiques d'aménagement, les SPLA. En effet, les opérations d'aménagement accessibles aux SPL sont les opérations visées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors que les SPLA « sont compétentes pour réaliser toute opération d'aménagement au sens du présent code », en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d'aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux SPL qu'aux SPLA la faculté de réaliser des opérations d'aménagement. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 octobre 2007, le second alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

d'ailleurs relevé dans votre intervention, monsieur Lefèvre. La mesure que vous proposez a des incidences juridiques qui dépassent largement la question de la définition des compétences des SPL, et qui n'ont manifestement pas été évaluées.

de cet amendement est d'élargir les compétences des SPL, sur le modèle de ce qui est prévu pour les SPLA, il serait alors préférable de cibler la mesure sur ce point

que les acteurs et les élus locaux puissent démontrer à l'administration, souvent encline à freiner les projets dans les départements ruraux, que le développement rural est inscrit dans la loi et qu'il n'y a pas de raison de s'y opposer systématiquement. Quel est l'avis de la commission J'entends la remarque tout à fait légitime de notre collègue Jacques Genest, mais je considère que les objectifs d'urbanisme déjà énumérés prennent largement en compte les enjeux ruraux, en citant notamment l'équilibre entre populations résidant dans les zones rurales et urbaines, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, ou encore la diversité des fonctions rurales et urbaines. Je ne suis pas sûre non plus du caractère normatif d'une telle mesure ... En conséquence, j'émets un avis défavorable

Malheureusement, il ne précise ni l'échéance ni le véhicule législatif. Celui-ci est pourtant tout trouvé, puisque le projet de loi que nous examinons en ce moment prévoit un certain nombre de mesures pour lutter contre l'étalement urbain. Il serait fort dommage de laisser passer cette occasion. Aussi, nous proposons de mettre en cohérence les objectifs du Gouvernement en inscrivant dans cette loi cette volonté d'arrêter l'artificialisation des sols, avec une échéance fixée à 2025. En effet, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. L'artificialisation du territoire est responsable de la perte de 236 hectares d'espaces naturels par jour, soit un département tous les sept ans ! Votre collègue Nicolas Hulot l'a parfaitement démontré, monsieur le ministre : l'urbanisation continue menace notre biodiversité. Toutes les espèces sauvages voient leurs habitats, quadrillés par nos routes et nos constructions, se réduire comme peau de chagrin. Au-delà des conséquences pour notre environnement, dont j'ai peur qu'elles ne suffisent pas, à elles seules, à vous convaincre, monsieur le ministre, arrêtons-nous un instant sur les conséquences sociales. L'étalement urbain entraîne une dégradation de la qualité de vie et de la santé des Français- allongement des temps de transport, pollution, etc. Ces phénomènes touchent, en premier lieu, nos concitoyens les plus démunis et entraînent un accroissement des coûts pour les collectivités territoriales. En effet, la diminution de la densité entraîne un renchérissement du coût des services publics- collecte des ordures, distribution d'eau potable, etc. Par ailleurs, l'urbanisation massive entraîne une aggravation des catastrophes naturelles, particulièrement les inondations. Le bétonnage massif réduit d'autant la capacité d'absorption de nos sols, aggrave les ruissellements et les conséquences des intempéries, intempéries, qui seront d'ailleurs amenées à se multiplier du fait du réchauffement climatique. Nous ne pouvons plus nous permettre de dégrader petit à petit notre environnement. Nous en sommes les principales victimes. Mes chers collègues, nous avons ici la possibilité d'agir et de respecter les engagements du Gouvernement.

saine, durable et accessible à tous, nous pouvons nous mettre d'accord sur cet objectif demandé par tous les syndicats agricoles. En effet, pour conserver la capacité de nourrir, demain, dix milliards d'êtres humains et pour préserver notre autonomie alimentaire, nous ne pouvons plus nous permettre de voir disparaître nos terres agricoles. Ce sont ainsi deux millions d'hectares qui ont disparu depuis trente ans, soit l'équivalent de la Gironde et des Landes cumulées, les deux plus grands départements français. Cette préservation des terres arables est d'autant plus indispensable que la détérioration de nos sols oblige à faire évoluer nos pratiques agricoles- alternance des cultures, développement du bio, etc. -, ce qui nécessitera davantage de surfaces agricoles utiles que notre actuel modèle intensif. Il est donc plus que temps de protéger les surfaces agricoles.

En complément des propos de notre collègue Guillaume Gontard, je précise que 58 % des constructions se font encore par artificialisation, laquelle est plus rapide que l'augmentation de la population. L'étalement urbain se poursuit, avec des conséquences non seulement sur les sols agricoles et la biodiversité, biodiversité, mais aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, ce phénomène s'accompagnant d'une augmentation du temps de trajet pour les ménages. Le Gouvernement a mis en place une feuille de route

dans le cadre du développement des territoires. Toutefois, le plan Biodiversité ne prévoit pas d'échéance, et je crois que 2025 est un horizon temporel nécessaire au regard de l'urgence de la situation.

doivent contribuer à atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2025. Quel

on ne peut pas légitimement interdire toute artificialisation, sous peine de porter un coup d'arrêt à la construction en zone rurale, et on voit mal comment la non-atteinte de l'objectif en 2025 serait sanctionnée. Et si cette mesure doit être considérée

Gouvernement ? Ces trois amendements visent à insérer l'objectif de zéro artificialisation nette dans les principes généraux de l'urbanisme.

dans lequel le ministre d'État, Nicolas Hulot, a souhaité qu'un groupe de travail soit mis en place, pour définir, en concertation avec les parties prenantes, l'horizon temporel à retenir pour atteindre cet objectif. J'en ai débattu avec Nicolas Hulot,

Saisi en 2016 par le ministère de la transition écologique et solidaire et celui des solidarités et de la santé, le HCSP a travaillé à l'identification des outils nécessaires à l'évaluation des impacts sur la santé dans les documents de planification territoriale relatifs aux déplacements, à l'urbanisme et au logement. Particulièrement attendu par les acteurs de terrain, le rapport comprend des recommandations structurantes, comme celle d'adapter le code de l'urbanisme de manière à prendre systématiquement en compte la santé au même titre que l'environnement, et des recommandations très opérationnelles pour favoriser l'utilisation d'outils d'intégration de la santé dans les trois documents de planification territoriale que chacun connaît.

Pour nous autres, Ultramarins, l'évocation de ces noms rappelle les ouragans récents, qui ont frappé nos territoires et causé des dégâts très importants, en plus des drames humains. Leur nombre et leur force ne cessent d'augmenter au fil du temps dix ouragans se sont ainsi succédé dans l'Atlantique entre août et octobre 2017. Ils sont la traduction du dérèglement climatique, qui affecte nos territoires au quotidien, comme le soulignait le rapport sénatorial d'information n° 131 de novembre 2015. a également des incidences sur des secteurs clés, tels que l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière, la pêche et l'aquaculture, ainsi que le tourisme. C'est pourquoi, s'il est reconnu en matière environnementale, le concept de résilience doit absolument être introduit dans notre politique de l'habitat. En effet, la résilience est la capacité de tout système urbain et de ses habitants à affronter les crises et leurs conséquences, tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne. une ville résiliente évaluera, planifiera et prendra des mesures pour se préparer et réagir à tous les aléas, qu'ils soient soudains ou à évolution lente, prévus ou non. Les villes résilientes seront donc mieux à même de protéger et d'améliorer la vie des citoyens. Pourquoi intégrer la résilience urbaine dans notre droit ? Tout simplement parce que, depuis 1992, le nombre de personnes touchées par une catastrophe est de 4,4 milliards, soit 64 % de la population mondiale, et les dommages économiques s'élèvent à environ 2 000 milliards de dollars. En 2015, quelque 117 pays et régions ont été frappés par une catastrophe. En conclusion, les gouvernements, les villes et les acteurs locaux doivent s'investir dans une démarche globale de résilience du logement social face à un risque majeur, penser de nouvelles modalités d'articulation entre développement urbain et prévention des risques et permettre, à terme, le développement d'une véritable culture sur le sujet dans les pratiques professionnelles du logement social. Le développement d'une telle démarche au sein du logement social des Antilles, démarche récompensée par le trophée de la résilience sociétale 2015, en est une bonne illustration. Bien sûr, les deux amendements que j'ai déposés sur ce sujet n'ont pas vocation

à M. Maurice Antiste. L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dresse un catalogue d'objectifs que doit viser l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme : équilibre entre populations résidant dans les zones urbaines et rurales, qualité urbaine, sécurité et salubrité publiques, prévention des risques naturels prévisibles, protection des milieux naturels ... Cet amendement vise à enrichir ce catalogue par une mention de la résilience, en particulier en particulier celle des constructions au changement climatique. En inscrivant la résilience à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, non seulement nous la consacrerions dans son principe en matière d'urbanisme, mais nous assurerions sa prise en compte, par ricochet, par un ensemble de documents de planification qui doivent s'attacher à respecter les objectifs de cet article. Il en irait ainsi

si chacune et chacun d'entre vous prend le soin de lire l'ensemble du code de l'urbanisme, vous verrez qu'il contient, en de nombreux endroits, plus d'incitations culturelles, disons des bonnes pratiques,

Il a vocation à répondre à l'urgence de la situation de tous les ménages qui attendent un logement social, faute de pouvoir se loger dans le parc privé. C'est une mesure emblématique du précédent quinquennat. L'enjeu est bien de construire des logements qui répondent aux besoins et aux revenus des Français. Il faut donc construire davantage de logements sociaux, en particulier dans les zones tendues. La construction de logements sociaux doit rester une priorité nationale. La cession des terrains publics contribuant à accélérer des opérations et à augmenter la capacité de financement du logement social. Elle est donc plus que jamais une nécessité. L'article 6 du projet de loi tend à abaisser le seuil de réalisation de logements dans les opérations réalisées sur du foncier public à 50 %. La cession des terrains de l'État représente un effort important de la Nation, qui doit continuer de favoriser essentiellement le logement. Le manque de foncier disponible et sa cherté sont suffisamment importants pour que la mobilisation des terrains de l'État soit orientée essentiellement soit orientée essentiellement vers le logement, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de consacrer une partie de l'opération à des commerces ou des activités autres, pour assurer une certaine mixité fonctionnelle. Le dispositif n'est peut-être pas parfait et pourrait encore être amélioré pour mieux atteindre ses objectifs, mais l'effet d'entraînement est indéniable : des opérations parfois bloquées depuis dix ans ont été engagées grâce à cette volonté politique affichée de produire plus de logements, notamment sociaux. Comment accepter que les terrains de l'État puissent servir des projets qui ne répondent pas à l'intérêt supérieur du pays ? Nous sommes donc très opposés au détournement de la vocation originelle du dispositif de cession du foncier public.

Le dispositif de décote Duflot permet à l'État de céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, en vue de la réalisation de programmes comportant « essentiellement des logements, avec une partie au moins de logements sociaux. Le projet de foi vient modifier le seuil des logements que doivent comporter ces programmes en l'abaissant à seulement 50 %, alors que le foncier public est rare et qu'il convient de ne surtout pas le brader. Aussi, la décote doit, à notre sens, être réservée uniquement à la relance de la construction de logements. Le présent amendement vise donc à préserver le taux de logements actuel au sein des programmes bénéficiant de la décote pour permettre de répondre aux besoins de nos concitoyens.

À l'inverse de ce projet de loi, qui porte comme seul avenir pour le patrimoine social sa vente à la découpe, nous militons pour la création d'un domaine public inaliénable. Notre proposition est simple. Il s'agit de renforcer les outils permettant d'agir de manière pérenne sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics accessibles.

Il s'agit d'abord de réaffirmer le rôle de l'État en matière de logement, donc de politique foncière. Il s'agit ensuite de sortir de la logique de fiscalisation de l'aide publique au logement et de renforcer l'aide directe de l'État à la construction, laquelle ne doit pas passer seulement par le subventionnement de la construction, mais aussi par les acquisitions foncières et immobilières directes nécessaires aux opérations publiques de construction de logements. Aujourd'hui, la Foncière est sous-dotée. Il faudrait revoir ses modes de financement. Nous souhaitons d'ailleurs, à l'instar de ce que propose le Gouvernement, que cette structure reste sous la responsabilité de l'État et non pas de la Caisse des dépôts et enfin de sortir les collectivités et opérateurs publics des difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui lorsqu'ils souhaitent participer à l'effort de construction, en reportant l'effort financier d'acquisition de terrains, qu'ils soient publics ou privés, sur cette agence. terrains appartenant à cette agence nationale foncière, les droits à construire ou à réhabiliter seraient confiés aux organismes HLM, pour produire des logements sociaux par un recours aux baux emphytéotiques à construction ou à réhabilitation. Les recettes liées à ces baux permettraient, à terme, à cette agence de s'autofinancer et, ainsi, d'engager le pays dans le cercle vertueux non pas de la diminution du parc social, mais bien de son essor. Concrètement, nous voulons faire évoluer le rôle de cette foncière vers l'acquisition de terrains ou d'immobilier afin de constituer un domaine public de l'État sanctuarisé, support de la production de logements sociaux et répondant donc à l'intérêt général. Voilà des pistes que nous estimons pertinentes et sur lesquelles nous souhaiterions que le Gouvernement travaille, pour faire de cette structure un acteur incontournable du logement public. L'amendement

Monsieur le président, cette conjonction de chiffres 7 ne peut que porter bonheur à cet excellent amendement. L'objet de cet amendement est de supprimer la mention d'une société codétenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que les prérogatives dérogatoires dont bénéficiait la Foncière publique solidaire pour permettre la réorientation de ses activités.

par l'article 50 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Cette société, codétenue par l'État et la Caisse des dépôts bénéficie de plusieurs prérogatives dérogatoires pour mener à bien sa mission de mobilisation du foncier public pour construire du logement, principalement social : un droit de préemption sur les cessions de foncier public ; un dispositif spécifique d'acquisition de gré à gré des terrains du domaine privé de l'État ; une application simplifiée de la décote, dont nous venons de parler ; des exemptions fiscales, telles que l'exonération des plus-values pour les tiers cédant des biens à la FPS, l'exemption de majoration de l'assiette de la taxe foncière ou l'exonération des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière. Depuis sa création effective, en mai 2017, cette foncière n'a pas pu développer ses activités, en raison des difficultés à monter rapidement des opérations importantes sur le domaine privé de l'État. Par ailleurs, il s'est révélé difficile de définir un modèle économiquement compatible avec l'exigence de construire une majorité de logements sociaux sur les fonciers acquis. Au travers de cet amendement, le Gouvernement souhaite réorienter le modèle de la FPS. La Caisse des La Caisse des dépôts et consignations va acquérir la totalité de ses parts, faire évoluer les missions de la société au service des bailleurs sociaux, avec un nouveau dispositif doté de 700 millions d'euros qui doit leur permettre

L'État peut céder des terrains relevant de son domaine privé à la Foncière solidaire s'ils sont destinés à la réalisation de programmes dont la majorité est constituée de logements sociaux. L'amendement du Gouvernement tend à supprimer cette obligation. C'est revenir complètement sur

de crédits qui pouvaient être disponibles pour de l'usufruit. Je voudrais être sûre que l'on n'entre pas dans des mécanismes qui ne seraient pas conformes à la tradition du logement social français. Qu'entendez-vous